La séance est reprise. Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, nous célébrons aujourd’hui la Journée internationale de la francophonie. Comme vous le savez, le Sénat a toujours apporté un soutien sans faille à la francophonie. Celle ci est d’abord une communauté linguistique, rassemblant plus de 320 millions de personnes. Au delà, elle est surtout une communauté humaine et culturelle, au sein de laquelle nos peuples ont tissé des liens profonds au fil du temps. La francophonie, c’est aussi, bien sûr, une communauté de principes, de valeurs telles que la paix, le dialogue, les droits humains et la tolérance, autant d’idéaux importants dans un monde contemporain traversé par la violence et les divisions géopolitiques, menacé par les extrémismes et fragilisé par la désinformation. Du 9 au 13 juillet prochain, le Sénat organisera, conjointement avec l’Assemblée nationale, la cinquantième session de l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF), en coordination étroite avec l’APF et sa section française. Il aura ainsi le plaisir et l’honneur d’accueillir les quelque 500 participants venant de tous les pays francophones qui sont attendus à ce grand événement. Mes chers collègues, Écologiste et Républicain, de la proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi n° 75 17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse,

nous pas des sujets exclusivement extérieurs et sans conséquence en France ? Certains pensaient même que modifier la Constitution en raison d’une menace lointaine et improbable, c’était surréagir. Depuis, J. D. Vance est venu à Munich expliquer aux Britanniques et, plus largement, à tous les Européens que les lois qui existent en Europe et qui sanctionnent le délit d’entrave à l’IVG étaient une atteinte à la liberté de conscience. Depuis, pour sa dernière soirée, la chaîne C8 a diffusé un film militant hostile à l’IVG. La menace anti choix a donc bien franchi, comme nous le craignions, les frontières des États Unis. Elle est même un objet d’ingérence du vice président américain et bénéficie de soutiens médiatiques et financiers colossaux. Notre proposition de loi s’inscrit dans la continuité de la loi Veil de 1975. Personne n’a, mieux que Simone Veil, dans une enceinte parlementaire, décrit le drame humain et sanitaire des avortements clandestins.

demandant la réhabilitation des femmes injustement condamnées, rappelant la souffrance de celles qui désiraient avorter avant 1975. Cette initiative a donné naissance à la présente proposition de loi, qui vise à prendre acte du préjudice subi par les personnes condamnées, et par toutes les femmes, avant la loi de 1975.

Depuis l’Antiquité, les États répriment l’avortement. Et les femmes continuent cependant d’avorter. Comme le dit très justement l’une des témoins du documentaire, du documentaire, une femme qui ne veut pas mener une grossesse à terme est prête à tout pour y parvenir, même à mettre sa vie en danger. Il en est ainsi depuis toujours.

Le code napoléonien poursuivait ainsi de travaux forcés les femmes qui avortaient. En 1892, les sanctions ont été aggravées et le corps médical s’est structuré autour d’une doctrine antiavortement. En 1920, les peines ont été encore renforcées et toute propagande anticonceptionnelle a été interdite. Pendant toutes ces années, on a toujours dénombré plusieurs centaines de milliers d’avortements clandestins par an. Sous le régime de Vichy, l’avortement devient un crime d’État et une femme fut même guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Dans l’immédiat après guerre, la peine de mort est certes abolie pour les crimes d’avortement, mais la répression est féroce.

Les deux guerres mondiales du XX siècle et leurs saignées démographiques sont suivies de politiques natalistes offensives : les femmes doivent repeupler la France et l’idée même du contrôle des naissances est fermement combattue.

Les hommes ont décidé seuls, aussi bien de la loi scientifique que de la loi politique. Leur seule connaissance de l’avortement était probablement celle qu’ils avaient des avortements de leurs maîtresses. D’ailleurs, leur lâcheté et leur hypocrisie leur épargnaient toute crise de conscience. La propagande antiavortement était fournie et dense., paru en 1943 et dédicacé par le maréchal Pétain, est à l’image de ce que l’on peut attendre de Vichy : la répression de l’avortement pour la défense de la race. En 1951, la République est revenue, mais le ministère de la santé publique et de la population publie. Nous relèverons la continuité des titres. Le substrat idéologique est différent, mais la conclusion est la même : il faut empêcher les femmes d’avorter et les peines doivent être dissuasives. pendant ces mêmes périodes, particulièrement au début du XX siècle, des femmes au courage insensé revendiquent le droit à la contraception et à l’avortement comme conditions de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je pense particulièrement à Nelly Roussel et à Madeleine Pelletier. Même au sein du mouvement féministe de leur époque, leur combat est précurseur. On peut et l’on doit aussi leur rendre hommage aujourd’hui. À partir des années 1950, et malgré la répression que j’ai évoquée, le mouvement en faveur du droit des femmes, du contrôle des naissances et du droit des femmes à disposer de leur corps commence à se structurer et à s’organiser.

la contraception (Mlac) et la méthode Karman, qui ont sécurisé les avortements clandestins, les cars vers l’Angleterre, l’inoubliable plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Marie Claire, le manifeste des 343 les manifestations féministes, pour qu’enfin l’avortement soit légalisé et pratiqué dans les hôpitaux. Il aura fallu tout cela pour qu’enfin on range les aiguilles à tricoter, les cintres, l’eau de javel, les décoctions de plantes toxiques et les cocktails de médicaments, pour qu’on en finisse avec les curetages à vif dans les hôpitaux « comme ça, ma petite fille, vous vous en souviendrez la prochaine fois ». Nous ne devons jamais oublier ni la violence du débat politique ni le courage de Simone Veil. Cette proposition de loi reconnaît que les lois antiavortement ont porté atteinte à la santé des femmes, entravé l’égalité, tué des centaines de milliers d’entre elles et en ont fait condamner des milliers. Elle reconnaît l’ensemble des souffrances que les femmes et leurs familles ont subies, y compris la honte à laquelle elles ont été assignées. Aujourd’hui, pour l’avortement comme pour le viol, la honte doit changer de camp. Parce que l’histoire des femmes et la place des femmes dans l’Histoire restent encore à écrire, cette proposition de loi installe également un comité chargé de recueillir les témoignages afin de documenter l’histoire des femmes qui ont connu l’avortement clandestin. Enfin, cette proposition de loi s’adresse aux millions de femmes auxquelles l’avortement est refusé et à celles qui luttent pour le défendre. Je la dédie aux 38 millions de femmes qui, chaque année sur la planète, sont contraintes de recourir à un avortement non sécurisé ou clandestin. Malgré l’offensive internationale, il y a des États qui ne plient pas. La France est de ceux là. En France, le consensus est solide. Il est renouvelé aujourd’hui et nous sommes déterminés. Aussi, je me réjouis de l’adoption imminente par le Sénat de cette proposition de loi. La parole

est il nécessaire que la loi reconnaisse la souffrance des femmes qui ont subi le drame de l’avortement clandestin avant la loi Veil du 17 janvier 1975 ? À cette question, la commission des lois a répondu positivement, et je souhaite vous expliquer pourquoi.

La souffrance des femmes du fait de l’avortement clandestin est incontestable. La présente proposition de loi nous offre simplement, dans son article 1, de la reconnaître officiellement, et c’est cette reconnaissance qui permet le travail de mémoire, en libérant la parole et en permettant le témoignage. J’ai été frappé par l’audition de Bibia Pavard, historienne et conseillère scientifique de la collecte de témoignages menée par l’Institut national

C’est parce que nous sommes là en dehors de toute démarche militante que la parole se libère et que la variété des situations – disons le, la variété des traumatismes – trouve à s’exprimer.

remplacé le terme « préjudice » par les termes « souffrances » et « traumatismes » afin d’éviter toute confusion. En effet, qui serait indemnisé ? Toutes celles qui ont souffert ? C’est évidemment impossible. Toutes celles qui ont été condamnées pour avoir subi un avortement clandestin ?

Pas plus qu’elle ne peut distinguer les bons et les méchants de l’Histoire, la loi ne peut choisir les « bonnes victimes Ce serait là un choix en décalage complet avec la volonté commune de faire face à la réalité historique de l’avortement clandestin. Dans son célèbre discours à la tribune de l’Assemblée nationale, la ministre de la santé d’alors, Simone Veil, montrait la nécessité de mettre fin

aujourd’hui, nous regardons en face notre propre histoire, une histoire de souffrances, d’injustices, mais aussi de courage et de détermination, une histoire de combats et de conquêtes, dans laquelle une chaîne ininterrompue de femmes a lutté sans relâche pour arracher à la morale et à la loi ce qui n’aurait jamais dû leur être confisqué : leur liberté, la liberté de maîtriser leur corps, la liberté de choisir leur destin. Oui, la République doit reconnaître. Oui, nous devons nous souvenir ; nous souvenir que, jusqu’en 1975, avorter pouvait être un crime. Entre 1870 et 1975, plus de 11 660 personnes ont été condamnées pour avoir avorté ou pour avoir aidé Sous Vichy, l’avortement devient même un crime à l’encontre de la sûreté de l’État et est passible de la peine capitale. Nous devons aussi nous souvenir de ces vies brisées par des grossesses non désirées, menées à terme sous la contrainte, dans la honte et le silence. Nous devons nous souvenir de celles qui ont tout risqué pour avorter dans la clandestinité. Il y avait celles qui arrivaient à prendre un car pour les Pays Bas ou un bateau pour l’Angleterre, mais à quel prix ? Il y avait celles qui se passaient en secret le nom d’un médecin qui pratiquait ces actes interdits. Il y avait surtout toutes celles qui ont eu à vivre les chambres sordides et les tables de cuisine, les cataplasmes brûlants, les aiguilles à tricoter, les cintres tordus, les fils de fer, les sondes de fortune. Il y avait celles qui mouraient.

Son avortement est comme ces milliers d’avortements clandestins, de ces avortements qui se passent mal, qui obligent à venir à l’hôpital en espérant être accueillie en urgence de ces avortements qu’on vous fait payer, puisqu’il fallait en plus faire souffrir ces jeunes filles, de ces avortements qui se finissaient avec des curetages sans anesthésie et qui laissent des traces indélébiles. Il y avait celles qui ne pouvaient plus jamais devenir mères, parce qu’il fallait bien expier la faute et qu’il y ait des conséquences. Il y avait celles qui étaient condamnées. Ménagères, secrétaires dactylos, vendeuses, institutrices, laborantines, ouvrières, étudiantes, ces femmes ainsi décrites par Gisèle Halimi, dans sa plaidoirie de 1972 de 1972 : « C’est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans argent et des sans relations qui est frappée. » Il y avait aussi celles et ceux qui les ont aidées : les médecins et les infirmières clandestins, les militantes, les mères, les sœurs, les filles, et ceux qui ont tendu la main. Madame la sénatrice, votre proposition de loi est un acte de justice envers ces milliers de vies brisées par des lois injustes et trop longtemps effacées de notre mémoire collective. Elle est un hommage à celles et ceux dont le courage a pavé notre chemin et que nous avons l’opportunité de réinscrire solennellement dans l’histoire des droits humains, dans l’histoire des droits des femmes. L’histoire de l’avortement, c’est l’histoire de nos mères, de nos grands mères, de toutes ces femmes anonymes qui ont refusé de plier. C’est l’histoire de générations de combattantes et de combattants, de militantes féministes et de citoyennes et de citoyens qui ont battu le pavé, défilé dans nos rues, exigé que les femmes puissent enfin décider pour elles mêmes. C’est l’histoire du manifeste des 343, ce coup de tonnerre du 5 avril 1971, lorsque des femmes, emmenées par Simone de Beauvoir, ont provoqué un débat inédit et forcé la société française à regarder en face sa propre hypocrisie. C’est l’histoire de Gisèle Halimi qui, en juillet 1971, fondait Choisir la cause des femmes et offrait sa défense aux femmes traquées par la justice pour avoir avorté, pour avoir repris le contrôle de leur propre C’est l’histoire du procès de Bobigny, à l’automne 1972, celle d’une adolescente de 16 ans, Marie Claire Chevalier, violée, dénoncée puis livrée aux tribunaux par son agresseur, celle de sa mère et de trois autres femmes, poursuivies pour l’avoir aidée. Et puis, il y eut ce jour du 17 janvier 1975. La France tournait enfin une page de honte et de silence. Ce jour là, la loi Veil entrait en vigueur, consacrant la dépénalisation de l’avortement. Cette victoire, si elle peut nous paraître évidente aujourd’hui, fut arrachée de haute lutte. Quelques semaines plus tôt, le 26 novembre 1974, Simone Veil montait à la tribune. Elle savait ce qui l’attendait : le mépris, les insultes, les attaques les plus ignobles, notamment antisémites. On tenta de l’humilier, de la faire plier, mais elle est restée debout, debout pour toutes celles qui n’étaient plus là pour témoigner, pour toutes celles dont la clandestinité avait marqué le corps, l’esprit et la réputation, pour toutes celles qui, sans cette loi, allaient encore risquer leur vie. Elle déclarait à la société tout entière que le temps des jugements, des peurs et des hypocrisies était révolu. Ces dernières semaines, nous avons célébré le cinquantième anniversaire de la loi Veil et le premier anniversaire de l’inscription, dans notre Constitution, de la liberté garantie des femmes de recourir à l’avortement. Cet acte était fort ; il était inédit. Et sans le Sénat, rien n’aurait été possible. Ce n’est certainement pas le point final de nos combats. C’est au contraire une déclaration : nous disons que la France est un pays où la dignité et la liberté des femmes sont des valeurs fondamentales, non négociables. La République ne transige pas avec les droits des femmes. La République ne transigera jamais avec la liberté des femmes. Et ce qui peut sembler être de l’Histoire ici ne l’est pas ailleurs. J’appartiens à une génération à qui l’on a appris que la marche de l’Histoire était une marche vers toujours plus de progrès, de droits et d’égalité. Nous avons grandi, peut être naïvement, en pensant que certaines conquêtes étaient irréversibles. Nous avions tort. Ce moment de bascule, où, comme le disait Simone de Beauvoir, « votre vie durant vous devrez demeurer vigilante », nous y sommes. Partout dans le monde, les droits humains, en particulier ceux des femmes, sont attaqués. Partout dans le monde, la liberté des femmes est contestée, fragilisée, éliminée. Partout dans le monde, les forces néoconservatrices, intégristes, islamistes, avancent. Partout dans le monde, et même à nos portes, elles n’ont jamais renoncé. Elles n’ont jamais désarmé. Elles guettent les failles, exploitent les crises, infiltrent les discours, opèrent des renversements, reviennent sur les libertés, détruisent des droits. Leur objectif est toujours le même : reprendre le contrôle des corps et des consciences. Ce sont non pas des menaces lointaines, mais des alertes. Alors oui, il nous faut demeurer vigilants. Et toute notre vie durant. Mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd’hui, nous avons la possibilité de réparer, mais surtout nous avons le devoir d’alerter. C’est pour cela que je vous appelle à voter cette proposition de loi le plus largement possible. Vous rendrez ainsi justice à celles qui ont combattu dans l’ombre, à celles qui ont payé de leur liberté, parfois de leur vie, le simple droit de disposer d’elles mêmes. Vous affirmerez ainsi une nouvelle fois haut et fort que la liberté des femmes n’a jamais été une concession. Elle a été, elle est et elle restera toujours une conquête, une conquête que nous devons protéger, une conquête que nous devons honorer, une conquête que nous devons transmettre, pour être à la hauteur de nos mères et de nos filles. La parole

il y a douze mois, nous étions réunis en Congrès pour inscrire dans la Constitution la liberté garantie à la femme de disposer de son corps. Cinquante personnes dans cet hémicycle s’étaient prononcées contre soit par opposition à la démarche, la trouvant inutile, soit par opposition à l’avortement, soit par refus que la France réagisse à une jurisprudence étrangère. Nous ne vivons pourtant pas sur une planète à part et devons bien prendre conscience du contexte international dans lequel nous inscrivons notre action. Je le répète régulièrement : ce que nous disons ici résonne au delà de nos frontières.

Nous étions une centaine de Français ; c’était inédit, et il était très important d’arriver en force. Dominique Vérien, présidente de la Délégation aux droits des femmes, m’a transmis l’extrait qui l’a le plus marquée dans la déclaration finale des États Unis Le gouvernement des États Unis n’encouragera plus les idéologies radicales qui remplacent les femmes par des hommes dans les espaces conçus pour les femmes Il ne dévastera pas non plus les familles en endoctrinant nos fils et nos filles pour qu’ils commencent à faire la guerre à leur propre corps, ou les uns aux autres. » Mes chers collègues, je n’avais pas conscience que défendre les droits de la moitié de l’humanité revenait à faire la guerre à l’autre… Ma famille n’a pas davantage conscience que, quand je cuisine pour elle, c’est une chance, et non une punition ! L’article 317 du code pénal, qui prévoyait une amende et une peine d’emprisonnement dans tous les cas d’IVG avant 1975, est resté en vigueur jusqu’en 2001 pour sanctionner les IVG ne respectant pas les conditions énoncées par la loi Veil de 1975. Anne Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, le rappelle : « Entre 1870 et 1975, 11 660 personnes ont été condamnées par l’État français pour avortement, aussi bien les femmes qui ont eu recours à l’IVG que les personnes qui les ont aidées. » Si l’on remonte encore dans le temps, un édit royal de février 1556 du roi Henri II exigeait que toutes les femmes célibataires ou veuves déclarent leur grossesse aux autorités. En l’absence de cette déclaration était créée une présomption d’infanticide en cas de perte de l’enfant à la naissance. Cette disposition digne du Moyen Âge existe encore dans certains pays. Mes chers collègues, si l’histoire de l’avortement nous enseigne bien une chose, c’est celle ci : les hommes légifèrent sur le corps des femmes depuis des siècles et dans tous les pays. Ces législations évoluent, pas toujours en bien, au gré des époques et des continents, mais une évidence persiste : le corps de la femme est un objet politique. Je tiens à cet égard à saluer l’engagement remarquable de notre collègue et auteure de cette proposition de loi, Laurence Rossignol, sur ces sujets. L’opportunité de ce texte est évidente, et je la remercie de l’avoir porté dans la Haute Assemblée.

visant à éviter dans le texte une ambiguïté pouvant conduire à un futur dédommagement financier des victimes de la politique anti IVG menée par la France. C’est un texte symbolique, donc, mais très important, car il contribue à un édifice encore fragile. La commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et traumatismes causés par les lois anti IVG, créée par l’article 2, sera dédiée au recueil de la parole, à la transmission des histoires tues et à la levée des tabous anciens. Elle offrira un lieu et un moment pour que notre société ouvre les yeux sur la réalité concrète et charnelle que nos lois imposaient encore récemment à la moitié de la population. Elle sera précieuse pour les générations qui nous ont précédés, mais aussi, et surtout, pour

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, un an après l’entrée du droit à l’IVG dans la Constitution et cinquante ans après sa légalisation par la loi Veil, nous reconnaissons aujourd’hui la souffrance physique et morale subie par les femmes ayant avorté en bravant l’interdit. Avec ce texte, la Nation admet que l’interdiction de l’IVG constituait une atteinte à la santé des femmes et à leur autonomie sexuelle et reproductive. Ce texte reconnaît la répression patriarcale exercée par l’État sur le corps des femmes. Nous saluons la création d’une commission nationale indépendante chargée de rétablir la vérité. Nous regrettons néanmoins l’impossibilité d’aller jusqu’à la compensation financière. Face à un État qui s’appropriait tous les droits sur le corps des femmes, celles ci ont dû longtemps se débrouiller seules. Avant 1975, l’avortement, c’étaient des pratiques dangereuses, parfois mortelles, causant des infections graves, des utérus transpercés, des hémorragies, des septicémies. Avant 1975, l’avortement, c’était risquer d’être traîné devant un tribunal, c’était s’exposer à des sanctions pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et à 100 000 francs d’amende. Sous le régime de Vichy, c’était même s’exposer à la peine de mort. Avant 1975, l’avortement clandestin, c’était la double transgression, à la fois sociale et pénale. C’était l’isolement, la stigmatisation, l’échec

L’écrivaine Annie Ernaux soulignait que « le paradoxe d’une loi juste est presque toujours d’obliger les anciennes victimes à se taire, au nom du “c’est fini tout ça”, si bien que le même silence qu’avant recouvre ce qui a eu lieu Avec cette proposition de loi, nous mettons fin à ce silence et nous reconnaissons la violence qui s’est exercée contre ces femmes innocentes. Les femmes ont payé de leur santé et de leur vie ce diktat sur leur propre corps. Avec ce texte, nous affirmons les coupables, ce ne sont pas les femmes qui avortent ni celles et ceux qui les ont aidées. Le coupable, c’est l’État, qui, en voulant contrôler le corps des femmes, les a mises en danger et les a condamnées. Rappelons que ce texte nécessaire arrive dans un contexte préoccupant de recul des droits sexuels et reproductifs : 47 000 femmes meurent chaque année des suites d’un avortement clandestin. Nous, parlementaires, avons constaté l’an dernier à quel point les mouvements antichoix étaient offensifs, financés et organisés. C’est une vérité : la désinformation prolifère et l’influence des assertions mensongères sur l’impact de l’avortement progressent chez les jeunes. En vérité, les femmes recourent à l’avortement à tout âge. Et à tout âge, recourir à un avortement, c’est risquer d’être confronté à un manque de compréhension de la part de certains professionnels de santé, à des jugements moraux et à des questions intrusives, stéréotypées ou culpabilisantes. Protéger le droit à l’IVG, c’est renforcer notre service public de santé, financer les centres de santé et les rendre accessibles partout en France. Ce texte nous renvoie aussi à notre haute responsabilité de continuer à lutter pour que le droit à l’IVG soit effectif. Le groupe CRCE K remercie l’auteure de cette proposition de loi. Nous sommes d’accord, il faut bien un devoir de mémoire. Notre responsabilité est d’écrire la vérité de l’histoire des droits des femmes, en commençant par recueillir la mémoire des atteintes à ces droits. Avec ce texte, la France regarde en face son passé. Nous voterons donc pour cette proposition de loi.

et de repentance dû aux millions de victimes qu’a causées la criminalisation de l’avortement en France. À toutes ces femmes, à toutes celles et à tous ceux qui les ont aidées, malgré les risques encourus, à maîtriser leur vie en ayant accès, clandestinement et donc dangereusement, à l’avortement, la France a envoyé un message puissant,

les cintres, les souffrances physiques, psychiques, sociales, économiques qui vous ont été infligées, nous n’aurions jamais dû les permettre et nous nous engageons, comme société, à ne plus jamais les accepter.

Lorsqu’une faute est établie, lorsqu’un préjudice est reconnu, cela entraîne des responsabilités. Cette responsabilité face aux victimes du passé s’étend aussi, politiquement, aux femmes d’aujourd’hui, à qui nous avons promis que leur liberté serait toujours garantie et qui peinent encore à accéder à ce droit fondamental

à bien des égards, nous rappelle les États Unis d’aujourd’hui. Le droit à l’avortement est partout attaqué par l’internationale réactionnaire, y compris en France, où les antichoix sont toujours là. Si nous Si nous reconnaissons notre responsabilité pour les victimes d’avant 1975, qu’avons nous à dire à celles qui meurent toujours en 2025 ? La responsabilité de la France, en votant cette loi, c’est bien de soutenir, face internationale réactionnaire, la solidarité féministe par delà les frontières, pour l’avancée des droits des femmes, et d’adresser un message puissant aux dizaines de millions de femmes toujours soumises aujourd’hui à la clandestinité.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et c’est heureux pour eux. Je vous parle d’un temps où la société patriarcale, l’ordre moral et le cadre légal envoyaient nos grands mères, nos mères, les épouses de certains d’entre vous peut être, devant les tribunaux, dans les cachots et même à l’échafaud. Je vous parle d’un temps où, en France, on entravait le corps des femmes. Je vous parle d’un temps où, en France, les femmes subissaient l’affront d’être jugées et condamnées, parce qu’elles avaient osé avorter. Je vous parle d’un temps où des femmes étaient contraintes d’avorter parce que le fruit de leurs amours ne répondait pas aux convenances sociales et aux attentes familiales. Je vous parle d’un temps où le troussage de domestiques, comme on le disait vulgairement, était monnaie courante, où le maître de maison engrossait la bonne avant de la mettre à la rue. Je vous parle d’un temps où les femmes, dans la nuit et le brouillard, montaient à bord de cars pour traverser la France et trouver un médecin compréhensif ou une faiseuse d’anges.

Je vous parle d’un temps où des militantes et des militants ont eu le courage de se lever et d’élever la voix. C’étaient les militantes du Mlac du MLF, c’était les « 343 salopes », c’était Gisèle Halimi, c’étaient ces victimes qui osaient témoigner à visage découvert lors du procès de Bobigny.

en participant à tous les mouvements émancipateurs pour les femmes dans notre pays et il a toujours été au rendez vous de l’Histoire. Aujourd’hui, en votant cette proposition de loi, nous adressons plusieurs messages. Nous disons tout d’abord aux femmes que la honte doit changer de camp. Aujourd’hui, en France, nous ne tolérerons plus qu’une femme soit obligée de baisser la tête, de mettre un genou à terre et de baisser les yeux tout simplement parce qu’elle a avorté.

le 26 novembre 1974, à la tribune de l’Assemblée nationale, Simone Veil présentait son projet de loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse. Elle s’exprimait en ces termes Personne n’a jamais contesté, et le ministre de la santé moins que quiconque, que l’avortement soit un échec, quand il n’est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Un demi siècle après la dépénalisation de l’avortement, nul ne saurait contester les souffrances, qu’elles soient physiques ou morales, endurées par ces femmes amenées à subir des avortements clandestins et par certaines des personnes y ayant procédé. Comment ne pas y être sensible ? Ce serait incompréhensible ! Réhabiliter la mémoire de toutes ces femmes condamnées pour avortement est un devoir. Si Simone Veil, en 1974, avançait que 300 000 femmes interrompaient leur grossesse chaque année, le nombre d’avortements clandestins ayant été pratiqués fait toujours l’objet de travaux de recherche, car il apparaît

celles de femmes qui, la plupart du temps, se sont trouvées seules à faire un choix impossible et qui ont finalement opté pour un avortement clandestin, à un prix souvent exorbitant et avec un risque très élevé de complications.

elle reconnaît les souffrances endurées aussi bien par les femmes ayant eu recours à l’IVG que par les personnes condamnées pour l’avoir pratiquée. elle institue une commission nationale indépendante auprès du Premier ministre, afin de collecter les témoignages des préjudices subis et transmettre la mémoire de ces derniers. Il s’agit bien d’un texte mémoriel, qui n’ouvrira aucun droit à des indemnisations ou compensations financières. La commission des lois a tenu à apporter cette précision, et je m’en réjouis. J’approuve également l’initiative de son rapporteur qui a modifié la composition de la commission nationale indépendante, en écartant les représentants de l’État et en y incluant des historiens et des chercheurs spécialistes du sujet. Madame la ministre, mes chers collègues, cinquante ans après la dépénalisation de l’avortement, il est primordial de réhabiliter la mémoire de toutes ces personnes qui ont subi, souvent au péril de leur vie, des avortements clandestins, ou qui les ont pratiqués. Alors que nous avons voté l’an passé, par la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse dans notre Constitution,

Désormais, l’interruption volontaire de grossesse est devenue un droit inaliénable, gravé dans notre texte suprême. Pourtant, alors que nous célébrons le cinquantième anniversaire de la loi Veil, réunis pour rappeler que ce droit n’a pas toujours été une évidence. Pendant plus d’un siècle, en France, avorter n’était pas seulement interdit : c’était un crime puni par la loi, réprimé par les tribunaux et combattu par la société. Des milliers de femmes ont été jugées, humiliées, privées de leur liberté, stigmatisées. Certaines ont tout perdu. D’autres y ont laissé leur vie. Aujourd’hui, nous avons un devoir : leur rendre justice. Tel est l’objet de cette proposition de loi, portée par ma collègue Laurence Rossignol, que je tiens à remercier. Elle vise à reconnaître officiellement l’injustice et les souffrances de ces femmes et à leur rendre leur dignité. Les conséquences de la législation répressive d’avant 1975 ont été dramatiques des centaines de milliers de femmes ont dû avorter clandestinement, dans des conditions souvent insoutenables, dans des arrière boutiques, sur des tables de cuisine, avec des aiguilles à tricoter. Elles ont subi l’infection, l’hémorragie, la peur et, parfois, la mort. L’État, par ses lois, n’a pas seulement bafoué la liberté des femmes ; il a aussi gravement mis en danger leur santé, au nom d’un puritanisme législatif. Les chiffres sont glaçants

seules, dans le silence absolu ? Nous avons inscrit la liberté de recourir à l’IVG dans la Constitution, afin de garantir à ce droit une protection supérieure. Mais comment pourrions nous prétendre défendre cette liberté sans reconnaître celles qui, avant nous, ont subi l’injustice ?

Je salue d’ailleurs l’excellent travail de la commission des lois et de son rapporteur Christophe André Frassa, qui a estimé incontestable la souffrance des femmes du fait de la législation antérieure à la loi Veil. créer une commission nationale indépendante chargée de recueillir leur parole, d’écrire leur histoire et de préserver leur mémoire, parce que cette dernière est un rempart contre l’oubli. Nous devons documenter ces récits, écouter ces femmes et leur redonner une voix. Il ne s’agit pas d’entamer une démarche indemnitaire ni de rouvrir des procès. Il s’agit d’un acte de vérité et de justice sociale. Il s’agit de dire, officiellement, que ces condamnations étaient une erreur. de loi, mes chers collègues, ne concerne pas seulement le passé. C’est un message pour l’avenir. Nous savons que les droits des femmes ne sont jamais acquis. Aux États Unis, en Pologne, en Hongrie, des gouvernements remettent en cause ce droit fondamental. Encore aujourd’hui, aux États Unis, des adolescentes sont contraintes de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un État où elles pourront avorter. Ne nous trompons pas : lorsque l’on cesse de défendre un droit, on prépare sa disparition. C’est pourquoi nous devons garantir un véritable accès à l’IVG sur tout tout le territoire français et assurer une vigilance constante. Réhabiliter ces femmes, c’est leur rendre justice, mais c’est aussi envoyer un message clair à toutes celles qui, aujourd’hui encore, doutent, culpabilisent, hésitent : votre liberté, mesdames, est légitime. Votre corps vous appartient, et jamais plus l’État ne doit vous le contester. Mes chers collègues, nous avons inscrit l’IVG dans la Constitution. Aujourd’hui, nous avons un autre devoir

nous sommes aujourd’hui réunis pour un moment de vérité, de mémoire et de justice. Il y a cinquante ans, la loi Veil reconnaissait aux femmes le droit de disposer de leur corps en dépénalisant l’interruption volontaire de grossesse. Mais avant cette date, avant cette victoire, la société et la République elles mêmes ont abandonné, condamné et brisé des milliers de femmes. Ces femmes n’étaient pas des criminelles. Elles étaient des mères, des sœurs, des filles, des amies. Elles étaient parfois trop jeunes, trop isolées, trop démunies. Elles étaient dans une détresse que nous ne pouvons qu’imaginer. Pourtant, elles ont été traquées, jugées, enfermées et, pour beaucoup d’entre elles, poussées à la clandestinité, au danger et parfois même à la mort.

En 1943, sous le régime de Vichy, une femme, Marie Louise Giraud, a été guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Autrement dit, elle a été exécutée pour avoir aidé d’autres femmes. Son nom restera à jamais comme le symbole d’une époque où la République a trahi ses propres valeurs et son humanisme. cinquante ans, une femme courageuse, Simone Veil, a brisé le silence de milliers de femmes pour lesquelles la liberté était non pas seulement une idée, mais aussi un droit. Elle s’est levée, telle une Marianne, pour briser l’omerta d’une souffrance qui, année après année, frappait des milliers de femmes.

L’histoire des femmes en France, c’est l’histoire d’un combat qui dure ; l’histoire d’une lutte permanente pour l’égalité, pour le droit de disposer librement de son corps, pour la liberté des femmes et leur place dans la société. Aujourd’hui encore, cette liberté est menacée. En Europe comme ailleurs dans le monde, des droits que l’on croyait acquis vacillent. Nous

refusons les antichoix. En adoptant cette proposition de loi, nous ne ferons pas qu’un acte de mémoire : nous accomplirons un acte politique. Réaffirmons le : la France ne tolérera jamais que l’on remette en cause la liberté des femmes. aujourd’hui : la République vous reconnaît, enfin. Et demain, nous continuerons à défendre le droit inaliénable des femmes à disposer de leur corps, sans peur, sans honte et sans jugement. La mémoire d’une nation reflète les valeurs d’une société. Sans mémoire, il n’y a pas de progrès. Sans transmission, il n’y a pas de justice. Changer le regard porté sur l’histoire des femmes, c’est refuser l’oubli. Changer le regard porté sur l’histoire des femmes, c’est défendre chaque jour la liberté de ces dernières. Changer le regard porté sur l’histoire des femmes, c’est bâtir collectivement l’avenir d’une société juste et

figurant au chapitre des crimes et délits contre les personnes, « quiconque aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte […] sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans Si l’avortement thérapeutique est finalement reconnu en 1852, la politique nataliste engagée dans les années 1920 durcit l’arsenal législatif. En la matière, le pic répressif est atteint sous le régime de Vichy, qui déclare l’avortement « crime contre la sûreté de l’État » et le rend passible de la peine de mort.

Je pense bien sûr à nos concitoyennes résidant à l’étranger, qu’elles vivent en Chine, en Arabie saoudite, au Maroc, au Sénégal ou encore aux Philippines. Pour elles comme pour les 750 millions de femmes qui, à travers le monde, vivent dans des États où le droit est restreint, voire bafoué, le combat pour les droits reproductifs et la liberté à disposer de son propre corps reste plein et entier, aujourd’hui, en 2025. C’est dans ce contexte global que s’inscrit, à mon sens, le présent texte,

l’histoire d’hommes qui se servent du corps des femmes, avec ou sans leur consentement ; l’histoire de la solitude des femmes, des retards de règles, des escaliers que l’on descend à toute vitesse, ou encore des tours de vélos que l’on fait toujours plus vite, en imaginant qu’ils permettront de se débarrasser d’une grossesse dont on ne veut pas.

Cette histoire, c’est la nôtre. C’est l’histoire qui nous a faites femmes et qui nous a faites féministes. C’est notre mémoire collective. Je me réjouis qu’elle devienne aujourd’hui une mémoire partagée et reconnue.

de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi n° 75 17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Victor Hugo disait : « Il est de règle que l’architecture d’un édifice soit adaptée à sa destination » – j’ajouterais à son environnement – « de telle façon que cette destination se dénonce d’elle même au seul aspect de l’édifice. »

rénovations, parfois désastreuses, contribuent à la standardisation de notre architecture, effaçant lentement les spécificités qui font la beauté de nos régions. Je sais que, dans cet hémicycle, nous dressons tous le même constat. Les travaux menés tant par Sabine Drexler que par Guillaume Gontard ont montré la nécessité de mieux protéger le bâti ancien et de soutenir la filière des matériaux biosourcés. Cette proposition de loi transversale lie des enjeux sociaux, environnementaux et culturels. Elle constitue un premier pas pour mieux protéger ce qui contribue depuis si longtemps à l’attractivité de la France. réhabilitation. Réhabiliter les bâtis anciens, c’est encourager une architecture, un urbanisme et un aménagement du territoire de qualité, respectueux de l’humain, de la nature et du patrimoine. Promouvoir la maison paysanne traditionnelle, réinvestir les centres villes anciens et les centres bourgs, c’est renouer avec des méthodes de construction plus écologiques. Avec cette proposition de loi pour une réhabilitation responsable du bâti ancien, nous souhaitons, à notre échelle, contribuer à réinventer un espace de vie collectif et durable, accessible à tous, concourant à créer les conditions d’une meilleure cohésion sociale. Le bâti ancien, dans sa conception bioclimatique, est résolument moderne. Sa réhabilitation et son entretien mettent à profit l’économie circulaire, l’artisanat et les ressources locales, ce qui contribue, ce faisant, au dynamisme de nos territoires. Mettre en valeur le déjà là, c’est promouvoir un logement qui vit avec son environnement en obtenant naturellement ce que l’on peine à reproduire artificiellement à grand renfort d’équipements énergivores. Le bâti ancien est innovant dans sa capacité à favoriser la circulation naturelle de l’air, à optimiser l’accès à la lumière, à bénéficier de la fraîcheur de la végétation comme de la chaleur de l’ensoleillement, et en réduisant les déperditions. C’est un mode constructif cohérent, favorable aux conforts d’été et d’hiver, tirant profit de l’inertie thermique de murs porteurs à la fois lourds et épais, de la régulation naturelle de l’humidité et de l’organisation intérieure des espaces.

majoritairement construits à l’aide de matériaux biosourcés, naturels et peu transformés, ayant parfois la propriété de stocker le carbone. Le bois, le torchis, le pisé, la terre crue, le roseau, le chanvre ou encore la paille sont ainsi parfaitement adaptés aux enjeux du bâti ancien. Ces matériaux se révèlent aussi performants que les isolants synthétiques ou minéraux. Privilégier ces isolants biosourcés permet d’éviter l’usage systématique de matériaux issus des énergies fossiles, dépendant de transports polluants et inadaptés à la rénovation des bâtis anciens. recouvrant de vieilles pierres d’un enduit en ciment, en apposant des plaques de polystyrène sur les murs ou en remplaçant des menuiseries en bois par des fenêtres en PVC, l’on provoque des dégâts irrémédiables.

Réhabiliter l’ancien, c’est œuvrer à la construction de logements durables, à une plus grande sobriété énergétique et à un meilleur confort pour les occupants. C’est aussi contribuer à un urbanisme circulaire, moyen tout à fait viable d’éviter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, en utilisant mieux l’existant.

Nous devons inciter l’État à soutenir financièrement les plus modestes, afin que le confort thermique ne soit plus un luxe et ne soit pas acquis au détriment des qualités et de la durée de vie du logement.

Mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur vous pour défendre cette modernité renouvelée, éclairée par la richesse de notre patrimoine bâti. La parole

également les conséquences néfastes d’une rénovation énergétique inadaptée au bâti ancien : celles ci sont esthétiques, culturelles, patrimoniales, mais aussi économiques et financières, puisque le soutien pécuniaire de l’État à la rénovation énergétique est vain s’il cible des travaux inadaptés.

Notre commission a donc salué l’initiative de notre collègue Michaël Weber, laquelle s’inscrit dans la lignée des constats et recommandations de Sabine Drexler, confirmés par ceux de la commission d’enquête sur l’efficacité

Je salue la qualité du dialogue et l’efficacité des échanges que j’ai eus avec Michaël Weber : cela nous a permis de parvenir à un accord sur le texte au stade de l’examen en commission.

À l’article 3, est mentionnée l’exigence de compétences supplémentaires spécifiques pour les auditeurs des bâtiments anciens, lorsque ces derniers présentent un intérêt patrimonial. En effet, même si des efforts ont été accomplis récemment, les connaissances des diagnostiqueurs sur les matériaux et les techniques traditionnels du bâti ancien sont bien souvent très insuffisantes.

Nous sommes en effet réunis aujourd’hui pour aborder un sujet crucial pour notre patrimoine et notre avenir : la rénovation énergétique du bâti ancien. Cette proposition de loi s’inscrit ainsi dans une démarche essentielle pour notre pays, visant à concilier la préservation de notre héritage architectural avec les impératifs de la transition énergétique et de la sauvegarde du pouvoir d’achat des ménages. Le bâti ancien, qui représente plus d’un tiers de notre parc immobilier, est un témoignage vivant de notre histoire et de notre savoir faire. Il est également un outil d’attractivité qui fait la richesse de nos territoires

si certains bâtiments anciens, grâce à l’usage de matériaux particuliers, sont très performants, d’autres sont de véritables passoires thermiques. Ainsi, en France, au 1 janvier 2024, quelque 29 % des résidences principales construites avant 1948 sont des passoires énergétiques classées F ou G selon le DPE, contre 14 % pour la moyenne des logements. Il nous faut donc rénover ces édifices, mais pas n’importe comment. la rénovation du bâti ancien présente des défis uniques, car les qualités intrinsèques, notamment hygrothermiques, des bâtiments concernés doivent être préservées. Une rénovation inadaptée peut non seulement réduire l’espérance de vie de ces bâtiments, mais aussi nuire au confort et à la santé de leurs résidents. une isolation thermique mal conçue, utilisant des matériaux inappropriés comme le polystyrène, peut provoquer une accumulation d’eau dans les murs, entraînant des pathologies pour les occupants. De même, le remplacement de fenêtres en bois, qui assurent une circulation essentielle de l’air et de l’humidité, par des fenêtres en PVC peut entraîner des effets de condensation et de moisissure. Ces exemples montrent l’importance de prendre en compte les spécificités du bâti ancien dans les projets de rénovation. Les ministères du logement et de la culture sont bien conscients de ces sujets, sur lesquels ils travaillent main dans la main. Ainsi, le Gouvernement a publié, la semaine dernière, un guide à l’attention des diagnostiqueurs immobiliers qui tend à mieux prendre en compte le bâti ancien dans le cadre du diagnostic de performance énergétique. Cette proposition de loi, déposée par le sénateur Michaël Weber, que je salue et remercie, vise à combler l’une des lacunes de la législation actuelle en adaptant certaines exigences de rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien.

Au sujet du DPE, permettez moi de rappeler que la ministre chargée du logement a lancé, cette semaine, un plan de dix mesures pour fiabiliser le diagnostic et lutter contre la fraude. Nous serons intraitables avec les diagnostiqueurs qui réalisent des DPE de complaisance et nous renforcerons la formation, notamment initiale, avec la création d’un cursus postbac. Je suis évidemment favorable à ce que cette formation intègre les techniques de rénovation du bâti ancien. Je ne puis terminer cette intervention sans évoquer le nerf de la guerre, à savoir les financements.

environnemental, pour garantir une rénovation durable et efficace. Le recours à ces matériaux favorise une économie locale qui concourt à la vitalité des territoires, tout en réactivant les savoir faire traditionnels. Ce sont d’ailleurs souvent les collectivités locales qui savent le mieux quel matériau employer ou quelle filière soutenir sur leur territoire. Comme ces matériaux coûtent plus cher, je vous annonce la parution, ce jour, d’un décret qui permettra aux collectivités de davantage financer le dispositif MaPrimeRénov’, en plus de l’aide nationale. Ce complément financera, notamment, des bonifications pour l’emploi de matériaux spécifiques, comme on le constate d’ores et déjà dans de nombreux territoires. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’examen de cette proposition de loi est l’occasion de montrer que la transition énergétique peut aller de pair avec la préservation de notre patrimoine. Ce texte est le fruit d’une réflexion approfondie et d’une volonté commune de trouver des solutions pragmatiques et équilibrées. En adaptant nos politiques de rénovation aux spécificités du bâti ancien, nous pouvons non seulement améliorer l’efficacité énergétique de notre parc immobilier, mais aussi préserver notre héritage culturel pour les générations futures.

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Nous débattons aujourd’hui des émissions de CO2 des logements et du bâti anciens, alors que le secteur du bâtiment est responsable de 25 % à 30 % des émissions de gaz à effet de serre.

la moitié des 15 millions de logements qui seront interdits en 2034 pourraient être considérés comme des bâtiments anciens. Cependant, faut il à ce titre les exonérer de rénovation et condamner à la précarité énergétique leurs résidents ? Certainement pas. Il est tout à fait nécessaire de soutenir la rénovation énergétique. Il nous faut mener cette bataille si nous voulons affronter les dangers du dérèglement climatique et des catastrophes qui en découlent. Nous en avons largement parlé lors des récentes inondations, et je crains que nous n’ayons, à l’avenir, besoin d’alerter encore

L’ancienneté des logements doit être prise en compte dans l’Hexagone, mais également en outre mer, y compris en intégrant les conditions climatiques particulières des collectivités concernées, comme celle de La Réunion. Tel est le sens de l’amendement du groupe CRCE K, qui sera présenté tout à l’heure. de loi va dans le bon sens, car il s’agit d’encourager tout le monde à rénover, y compris lorsque c’est difficile, lorsque le bâti est spécifique. Or c’est le cas pour les logements construits il y a un siècle. Cependant, les difficultés techniques trouvent souvent des réponses économiques, dès lors que nous nous en donnons les moyens – je vous ai bien entendu, monsieur le ministre… À ce titre, je regrette que les subventions supplémentaires

l’équation est claire : construire un immeuble nécessite soixante dix fois plus de matériaux et produit cinq fois plus d’émissions de gaz à effet de serre qu’une réhabilitation. Les rendez vous du siècle nous imposent donc de ne démolir qu’en dernière extrémité, de focaliser nos efforts sur la transformation de l’existant et de construire moins, beaucoup

L’enjeu est donc immense. Il nécessite la mobilisation des savoirs et des matériaux que le simplisme du béton avait jusqu’à récemment effacés de nos mémoires et de nos chantiers. Les bâtiments anciens sont le reflet de l’identité et du patrimoine de nos régions, comme Michaël Weber l’a bien rappelé. Ils doivent être préservés et rénovés en respectant nos savoir faire autant que l’environnement, grâce à l’utilisation de matériaux bio et géosourcés, dont ils sont composés à 90 %.

de près de 100 % depuis quatre ans. Rappelons encore que ces matériaux durables ne sont pas uniquement prédisposés à la rénovation de l’ancien et progressent aussi beaucoup dans le neuf.

La rénovation thermique des bâtiments est le chantier du siècle. Elle devrait d’ailleurs être incluse dans la stratégie de sécurité globale de notre pays. Souveraineté énergétique, décarbonation de l’économie, artisanat et économie des territoires, ainsi que, évidemment, pouvoir d’achat, confort et habitabilité des logements hiver comme été

l’histoire des lieux et ce qui nous lie aux autres générations. Les lieux fabriquent des liens qui permettent de créer ensemble une société plus solidaire et conviviale. » La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2021, nous ne cessons de rectifier, de préciser et de corriger les écueils et mesures inapplicables de la loi Climat et Résilience. La semaine dernière, nous examinions la

fixer des objectifs ambitieux est impératif, mais se donner les moyens de les atteindre l’est tout autant. Soyons clairs : il est indispensable de réduire les répercussions des bâtiments sur l’environnement. Nous devons

Comment pouvons nous, en effet, évaluer la performance énergétique d’un édifice datant du début du siècle dernier avec la même grille d’évaluation que celle qui est utilisée pour des constructions récentes ? Tout cela est insensé. Pourquoi inciter à des rénovations utilisant des méthodes d’isolation modernes, inadaptées au bâti ancien ? Cette approche nous pousse à privilégier des matériaux qui présentent un un impact environnemental fort et qui dénaturent notre patrimoine. C’est pourquoi cette proposition de loi, qui tend à prendre en compte les spécificités du bâti ancien, est parfaitement judicieuse. Nous nous réjouissons des ajouts opérés par Mme la rapporteure, notamment la nécessaire prise en compte des spécificités thermiques du bâti ancien dans le diagnostic de performance énergétique. Il est en effet indispensable de considérer ses atouts, notamment

Par ailleurs, nous devons aussi simplifier. Ainsi, restaurer un édifice ancien suppose des connaissances spécifiques : il convient de connaître les savoir faire et les matériaux traditionnels. Faut il, cependant, mobiliser un architecte des Bâtiments de France (ABF) pour chaque audit ? Personnellement, je ne le crois pas.

tous les bâtis ne se valent pas. Aussi, nous soutenons que c’est uniquement lorsque ces édifices présentent un fort intérêt patrimonial qu’il est souhaitable de faire appel à l’auditeur. Là non plus, ne tombons pas dans une rigidité excessive, laquelle, pour régler un problème, en créerait un autre

qui illustre de manière édifiante la menace qui pèse aujourd’hui sur le patrimoine bâti ancien en France. Sa situation est symptomatique d’une tendance préoccupante, qui sera largement évoquée lors de nos débats : la difficulté à concilier préservation du patrimoine, enjeux économiques, réglementations actuelles et transition énergétique. Ainsi, en novembre 2022, une maison du XVI siècle, recouverte de crépi et affublée d’annexes, d’annexes, qui n’avait plus l’air de rien, ou presque, devait être démolie pour permettre la réalisation d’un lotissement. Cependant, elle a été sauvée grâce à la vigilance de deux passionnés d’architecture rurale, l’inspection clandestine a révélé, sous le crépi et à l’arrière des annexes, une structure en pan de bois datant de 1554, caractérisée par des éléments architecturaux remarquables et des bois de forte section en parfait état. Face à l’urgence de la situation, une mobilisation citoyenne s’est rapidement organisée, et suffisamment de fonds ont été collectés pour procéder au démontage méthodique de la maison avant le jour programmé de sa démolition. Elle sera très prochainement remontée au Parc de la Maison alsacienne à Reichstett, dans le Bas Rhin, offrant ainsi une perspective sur l’architecture alsacienne du XVI siècle. Cette initiative met en exergue l’importance de la vigilance et de la mobilisation collectives pour la sauvegarde du patrimoine architectural de nos régions.

ou dans des écomusées, car leur vraie place est là où elles ont été construites. L’Alsace est une région reconnue pour ses maisons traditionnelles, qui font partie de son identité culturelle et attirent, chaque année, des millions de touristes. Pourtant, 300 d’entre elles disparaissent chaque année, soit par démolition, comme ce qui a failli arriver à Buschwiller, soit à la suite de rénovations inappropriées, qui portent atteinte à leur structure au point de les condamner quelques années plus tard à la démolition. Ce phénomène s’est encore accéléré avec la loi Climat et Résilience, dont nous mesurons tous qu’elle a des effets pervers qui n’ont pas été anticipés.

en valorisant les métiers du patrimoine et en développant les formations qui permettent de les exercer, mais aussi en encourageant les communes à identifier et à protéger leur patrimoine bâti. À cette fin, sensibiliser les habitants

Le bâti traditionnel incarne une intelligence constructive, dont nous devons désormais nous inspirer. À nous donc de faire de la transition énergétique une chance.

en matière de rénovation énergétique, présidée par Dominique Estrosi Sassone, soient aujourd’hui débattues. Je ne doute pas que, ensemble, nous réussirons à faire progresser notre législation, certes à petits pas, mais dans le bon sens. Je salue

la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à concilier performance énergétique et préservation du bâti ancien, un enjeu central de notre transition écologique et de la valorisation de notre patrimoine architectural. Je tiens à saluer l’initiative de notre collègue Michaël Weber, ainsi que le travail approfondi mené par la commission des affaires économiques. Je remercie également Mme la rapporteure, Sylviane Noël,

il est également un défi de taille en matière de rénovation énergétique, car il ne saurait être traité comme le bâti plus récent. Nous avons collectivement affirmé notre engagement pour la transition énergétique au travers de la loi Climat et Résilience de 2021. Toutefois, force est de constater que les spécificités du bâti antérieur à 1948 ont été insuffisamment prises en compte dans les dispositifs de rénovation, comme l’a souligné la commission d’enquête sénatoriale relative à l’efficacité des politiques publiques en la matière. Il est donc impératif d’adapter nos outils et nos méthodes aux réalités du terrain. Aujourd’hui, de nombreux propriétaires de bâtiments anciens sont confrontés à des injonctions contradictoires et subissent des obligations de rénovation qui ne tiennent pas compte des caractéristiques techniques et patrimoniales de leurs biens. sont mal calibrées, voire inadaptées. Ce constat appelle donc des ajustements législatifs. C’est sur ce point que cette proposition de loi est particulièrement importante et pertinente : elle porte des avancées majeures, à commencer par l’inscription des définitions

Enfin, nous devons accorder une attention particulière aux territoires ultramarins, dans lesquels les spécificités climatiques et architecturales imposent des approches sur mesure. La réglementation thermique, acoustique et d’aération de 2010 a permis des avancées, notamment en favorisant la ventilation naturelle pour limiter l’usage de la climatisation. Ce type d’adaptation doit inspirer notre approche du bâti ancien dans son ensemble. Le groupe RDPI RDPI soutiendra donc ce texte pragmatique et utile pour les rénovations de nos bâtis anciens. La parole

représente un tiers du parc de logement pour 39 % de sa consommation d’énergie. Ses performances en la matière en font donc un gisement important d’économies d’énergie, ainsi qu’un levier non négligeable de lutte contre la précarité énergétique. Pourtant, les outils mis à disposition par le législateur en matière de rénovation énergétique sont uniformes pour l’ensemble des types de bâtis et se révèlent donc inadaptés au bâti ancien, au point de menacer sa préservation.

Ce n’est qu’en conciliant tous ces paramètres que l’on préservera ses qualités historiques, architecturales, techniques, ses performances intrinsèques et son confort en été comme en hiver. Nous devons veiller à ne pas créer de déséquilibres et prendre impérativement en considération le fait qu’il relève d’un système constructif particulier, vernaculaire, ayant recours à des matériaux naturels locaux et peu transformés, à base de pierres, de bois ou de terre cuite ou crue. C’est pourquoi ce texte, en faisant évoluer le DPE pour tenir enfin compte des qualités constructives du bâti ancien, notamment de ses spécificités thermiques et des caractéristiques hygrothermiques des matériaux le composant, constitue un pas nécessaire vers une transition plus juste. Il y va tout simplement de l’acceptabilité d’une politique souhaitable, mais qui, pour réussir, exige d’être comprise et non contestée en raison des exigences issues de sa mise en œuvre. Soyons vigilants à ne pas laisser notre volonté de répondre de manière rapide et massive aux défis posés par l’urgence climatique nous conduire dans une impasse, d’autant que le bâtiment ancien, souvent dégradé, est occupé majoritairement par des publics précaires. S’il n’est pas question de contester le bien fondé du DPE ni les contraintes, voire les sanctions, imposées aux logements identifiés comme des passoires thermiques, ce système nécessite une adaptation au bâti ancien.

Ce phénomène d’éviction du logement locatif permanent, déjà présent dans certaines communes, constitue une source d’injustice pour les milliers de Français bloqués dans leur parcours résidentiel, mettant à mal le pacte social et menaçant la solidarité et la cohésion nationale.

C’est pourquoi, pour lutter contre la désertification programmée de nos centres bourgs et de nos villes, où se trouvent la plupart des habitats anciens, et contre la disparition d’une partie de notre patrimoine par la perte de savoir faire, il est nécessaire de mieux concilier les objectifs de la rénovation thermique avec ceux

Nous serons ainsi particulièrement attentifs aux différentes solutions que proposera le rapport. Le soutien financier aux travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens est en effet indispensable pour les ménages les plus modestes, donc essentiel pour son acceptabilité.

la rénovation énergétique des logements s’est progressivement imposée comme une politique publique essentielle située au carrefour des différents défis auxquels nous devons faire Tout d’abord, elle répond à un enjeu environnemental, dans la mesure où le bâtiment constitue le troisième secteur d’émissions de gaz à effet de serre, avec 18 % des émissions nationales et 45 % de la consommation finale énergétique. Ensuite, elle répond à un enjeu social, dans un pays où 30 % des ménages ont souffert du froid en 2023, au sein des 5,2 millions de logements considérés comme énergivores. Enfin, elle répond à un enjeu économique, dans un contexte où nous devons repenser notre modèle d’aménagement des territoires. En effet, si 80 % des logements de 2050 existent déjà, les deux tiers d’entre eux sont mal isolés. Alors que les surfaces constructibles deviennent de plus en plus rares, le dérèglement climatique et la dévitalisation des centres bourgs nous imposent de mener une politique plus rigoureuse en matière de rénovation, y compris énergétique. À de multiples reprises, et de plus en plus fréquemment, le législateur s’est interrogé sur l’orientation sur l’ambition à donner à cette politique. Qu’il s’agisse d’accélérer, d’assouplir ou de supprimer le calendrier de rénovation des passoires thermiques, voire de donner des marges de manœuvre aux acteurs publics ou privés pour atteindre les objectifs, les normes législatives et réglementaires en la matière fluctuent en fonction des crises, alors que le secteur du bâtiment demande de la stabilité et de la simplification. C’est dans ce contexte qu’un rapport d’information de la commission de la culture sur le patrimoine et la transition écologique a conclu, en juin 2023, que la législation actuelle ne tenait pas suffisamment compte des qualités du bâti ancien, à l’exception des bâtiments historiques. La présente proposition de loi découle de ce travail. Elle aborde le cas du bâti ancien, une catégorie regroupant les bâtiments achevés avant 1948, qui représente un tiers de notre parc national. Ce type de bâtiment est singulier : il est composé de matériaux naturels et exige une réhabilitation spécifique, incompatible avec les techniques et les matériaux utilisés sur le bâti moderne. Autrement dit, le bâti ancien nécessite des procédés de réhabilitation rigoureux et individualisés, afin d’améliorer la performance énergétique des lieux, tout en conservant ses qualités intrinsèques et sa valeur patrimoniale. Tels sont les principaux objectifs de cette proposition de loi. Pour y répondre, ce texte propose d’inscrire dans le marbre la définition de bâtiment ancien, qui se caractérise par une faible empreinte environnementale.

nions pas le rôle de la défiance des particuliers envers certains indicateurs et outils complexes, comme le DPE et le RGE, comme frein au déclenchement des travaux. Et je n’aborde même pas le reste à charge, qui représente en moyenne 65 % des dépenses engagées. Cette proposition de loi adapte également les modalités de l’audit énergétique aux bâtiments anciens, en imposant que les propositions de travaux soient adaptées aux contraintes architecturales et patrimoniales pesant sur l’édifice Cette exigence se double d’une attente de compétences supplémentaires spécifiques au bâti ancien. Cette dernière mesure est alignée avec l’impératif d’un vaste plan national et ambitieux de formation à la rénovation énergétique des logements,

Au delà de la problématique du reste à charge, cette question doit être abordée de manière plus large et ambitieuse. L’idée d’une planification pluriannuelle pourrait ainsi être expertisée afin de donner des perspectives budgétaires à toute la filière, laquelle pourrait alors monter en puissance et en compétences.

En définitive, cette proposition de loi nécessaire repose sur deux fondements. D’une part, elle répond aux problématiques posées par le poids du bâti ancien dans le parc de logements et par les singularités des réhabilitations à y effectuer ; d’autre part, elle nous rappelle les multiples défis qui jalonnent notre politique, tels que la formation, la simplification et le financement. Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte.

nous examinons aujourd’hui une proposition de loi essentielle, déposée par notre collègue Mikael Weber, sénateur de la Moselle, qui vise à adapter les enjeux de la rénovation énergétique de la rénovation énergétique aux spécificités du bâti ancien. La rénovation énergétique est une priorité nationale. Nous voulons tous réduire la précarité énergétique, limiter l’artificialisation des sols et atteindre nos objectifs climatiques, mais ces ambitions doivent tenir compte des réalités du bâti existant. Or la législation actuelle est mal adaptée aux bâtiments anciens, qui représentent plus d’un tiers du parc immobilier. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 repose sur des critères pensés pensés pour le neuf et ignorant les spécificités des constructions d’avant 1948, avec pour résultat des obligations de travaux inadaptés, voire nuisibles. Prenons un exemple. Une maison en pierre du XIX siècle, typique des centres villes et des campagnes, a été conçue avec des matériaux respirants comme la pierre, la chaux et le bois. Son isolation repose sur un équilibre hygrométrique naturel. Pourtant, les normes en vigueur imposent souvent une isolation intérieure avec des matériaux étanches comme le polystyrène ou la laine de verre. qui, auparavant, circulait librement se retrouve piégée, entraînant moisissures, condensation et dégradations structurelles. Pis encore, des travaux inadaptés sont souvent exigés pour que ces logements restent louables. Des propriétaires bien intentionnés, mais mal accompagnés, en viennent ainsi à financer des rénovations qui accélèrent la détérioration de leurs biens au lieu de l’améliorer. À cela s’ajoute un autre problème essentiel : le manque de soutien financier adapté. Les aides comme MaPrimeRénov’ sont souvent inaccessibles ou mal calibrées pour le bâti ancien ; les dossiers sont complexes, les délais longs et les montants incertains, rendant les rénovations coûteuses et risquées. Les matériaux compatibles avec les constructions anciennes sont souvent plus chers, mais, paradoxalement, moins bien subventionnés que des solutions inadaptées. Les propriétaires de maisons anciennes en souffrent particulièrement. Faute d’aide adaptée, nombre d’entre eux doivent vendre ou abandonner des biens qu’ils auraient voulu préserver. Cette situation est préoccupante. Nous risquons de voir disparaître un pan entier de notre patrimoine, faute de solutions viables pour le rénover. Il est donc urgent d’adopter une approche plus rationnelle et plus respectueuse du bâti ancien. La proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui s’articule précisément autour de plusieurs axes visant à adapter les critères d’évaluation énergétique aux spécificités des bâtiments anciens. Elle modifie l’audit énergétique, qui devient un audit énergétique et patrimonial réalisé par des professionnels spécialisés ; elle encourage l’utilisation de matériaux compatibles, en renforçant les aides financières pour les matériaux biosourcés et géosourcés, respectant les propriétés physiques des bâtiments anciens ; enfin, elle garantit une rénovation saine en imposant une vigilance accrue sur la gestion de la ventilation et de l’hygrométrie, afin d’éviter les effets délétères d’une isolation inadaptée. Cette proposition de loi vise non pas à freiner la modernisation de notre parc immobilier, mais à la rendre plus intelligente et plus respectueuse des réalités architecturales comme des techniques du bâti ancien. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à la voter sans hésitation.

cette proposition de loi de mon collègue Michael Weber s’inscrit dans la continuité de la priorité que s’est fixée le groupe socialiste : donner une importance considérable à la question de la rénovation thermique des bâtiments. Après la proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique, que j’avais eu l’honneur de défendre devant vous, après le texte portant sur l’adaptation des matériaux et des normes de construction aux spécificités et aux contraintes des outre mer de ma collègue Audrey Bélim,

Il fait la fierté de nos territoires, de nos communes. Il est la traduction de l’intelligence et de l’ingénierie de ceux qui nous ont précédés. Ceux ci ont su concevoir des bâtiments vivants, optimisant les bénéfices de leur environnement proche tout en réduisant ses inconvénients. Le bâti Le bâti ancien vit avec son environnement grâce à un équilibre subtil et fragile que nous devons préserver. Il est le fruit

Il s’agit de la maison en pan de bois et en torchis blanchi, chez moi, dans la Somme, du mas de Provence, de la chaumière normande ou de la maison basque. Parce que la France est un pays riche de ses terroirs, le bâti ancien est infiniment varié. varié. Il se caractérise par le recours à des méthodes de construction vernaculaires et à des matériaux naturels peu transformés et d’origine locale, tels que la pierre

a été conçu pour s’adapter à son environnement. Vous l’aurez compris, l’ambition de cette proposition de loi est de préserver notre habitat ancien et sa qualité architecturale, en contribuant à améliorer ses performances énergétiques. Le bâti ancien représente environ 11 millions de logements, soit un tiers du parc français. 70 % du bâti construit avant 1948 sont classés F, E ou G, c’est à dire dans la catégorie des passoires thermiques. Alors que la France s’est engagée à diminuer de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre et de 30 % sa consommation d’énergie fossile à l’horizon de 2030, la rénovation thermique joue un rôle central dans la lutte contre le dérèglement climatique. La rénovation du bâti ancien est donc primordiale pour remplir nos objectifs en matière d’engagement écologique, mais aussi pour améliorer le confort de vie d’un certain nombre de nos concitoyens. Il s’agit enfin d’un enjeu de justice sociale : éradiquer les passoires thermiques

Une rénovation inadaptée, appuyée sur des techniques et des matériaux contemporains peut causer des désordres, comme la perte de la régulation naturelle de la température et du taux d’humidité, diminuant l’espérance de vie du bâti et nuisant au confort de vie et à la santé de ses occupants. La rénovation du bâti ancien offre également une promesse d’avenir. En plus de leur valeur patrimoniale, qui contribue à la richesse et à l’identité de nos régions, les bâtiments anciens offrent des avantages majeurs pour faire face au réchauffement climatique grâce à une faible empreinte environnementale et à une empreinte carbone déjà amortie.

ainsi que les matériaux biosourcés réduisent nos dépendances aux importations et diminuent l’empreinte carbone des produits, favorisant à la fois l’économie locale et la souveraineté industrielle, en valorisant les ressources disponibles sur nos territoires. La rénovation du bâti ancien, particulièrement en milieu rural, joue un rôle clé dans la lutte contre l’artificialisation des sols et pour la revitalisation de nos centres bourgs. Pour préserver ces centres historiques, il est essentiel que ceux ci restent habités. Par ailleurs, combattre la précarité énergétique offre un levier pour redynamiser ces espaces. Cette démarche soutient également les filières artisanales, en valorisant des savoir faire transmissibles, des formations et des emplois locaux non délocalisables. Notre bâti ancien mérite donc

des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments anciens à usage d’habitation. Mes chers collègues, voter cette proposition de loi, c’est faire preuve de pragmatisme. C’est renouer avec l’intelligence, l’ingénierie et le savoir faire des artisans de nos territoires. C’est contribuer à améliorer près de 11 millions de logements, soit un tiers du parc français. C’est préserver et valoriser notre histoire,

La réhabilitation, telle qu’elle est définie dans le droit européen, n’existe pas dans notre code de la construction et de l’habitation, alors qu’elle est largement utilisée par les personnes travaillant dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel matériel. Alors que la rénovation peut être plus intrusive et transformer significativement un bâtiment, sans nécessairement respecter son matériau ou son intérêt patrimonial, la réhabilitation est une démarche plus respectueuse du bâti existant, qui vise à conserver et à valoriser les éléments d’origine, tout en les adaptant aux normes modernes. Elle est, pour cette raison, souvent utilisée pour des bâtiments patrimoniaux, avec l’objectif de préserver l’authenticité et l’identité architecturale tout en améliorant le confort et la sécurité. Cet amendement

de remplacer la notion de rénovation énergétique du bâti ancien par celle de réhabilitation du bâti ancien. MaPrimeRénov’, par exemple, est destinée à financer la rénovation énergétique, et non la réhabilitation.

conclusions du rapport de la commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation thermique. Ces matières premières présentent de très nombreuses qualités, parmi lesquelles le

Par ailleurs, la filière française de matériaux d’isolation s’appuie aujourd’hui largement sur des produits d’isolation géosourcés et biosourcés fabriqués en circuit court à partir de matières premières locales renouvelables, notamment issues de l’agriculture, comme la paille et le chanvre.

des matériaux biosourcés et géosourcés, mais on ne soutient pas une filière en introduisant des définitions dans la loi ! La commission des affaires économiques a supprimé ces définitions non par opposition à ces matériaux, mais parce qu’elles risquaient d’être trop restrictives et inadaptées. Par exemple, le ciment aurait pu figurer dans la liste des matériaux géosourcés…

car toutes les problématiques auxquelles le bâti traditionnel est aujourd’hui exposé sont liées à l’absence de protection ou, tout du moins, d’identification, tout particulièrement dans la ruralité,

nette (ZAN) et du DPE –, il est aujourd’hui plus qu’urgent d’inciter les élus locaux de notre pays à répertorier leur bâti patrimonial dans les documents d’urbanisme, afin de limiter les travaux inappropriés et, à terme, d’éviter d’ailleurs ce qui se fait dans ma région, la Collectivité européenne d’Alsace ayant mis en place un dispositif qui majore les subventions accordées en cas de travaux de réhabilitation sur le bâti non protégé lorsque les collectivités locales ont procédé à cette identification et à son inscription dans les documents d’urbanisme. C’est une politique qui, je le précise, rencontre un très grand succès.

environnemental des matériaux et intègre et favorise l’emploi de matériaux biosourcés et géosourcés, plus écologiques. De fait, en tenant

Aujourd’hui, nous constatons tous que la réglementation du DPE est inaboutie et que des adaptations sont nécessaires, notamment pour le bâti ancien, qui représente plus de 30 % des logements.

la simplification normative et la lisibilité, pour que nos concitoyens gardent confiance dans le DPE et pour que les professionnels puissent rester mobilisés. Il y a déjà eu deux réformes du DPE. Je rappelle que la prise en compte du confort d’été est satisfaite par l’article 1, dans sa rédaction issue des travaux de la commission. Le renouvellement de l’air

une rénovation énergétique performante. Cette mesure va bien au delà de la seule prise en considération des spécificités du bâti ancien dans les obligations de rénovation énergétique.

s’appliquant à la fois à la construction, à la rénovation et à l’entretien des bâtiments et prenant en compte divers critères. Sur ce point, l’amendement est déjà satisfait sur le fond : de telles et de l’habitation, qui fixe des exigences multicritères pour la construction et la rénovation des bâtiments. L’amendement n° 23 a également pour objet que la réglementation thermique établisse des règles spécifiques

Enfin, cet amendement tend à privilégier l’utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés dans la rénovation des bâtiments anciens. Or le choix des matériaux doit pouvoir se faire au cas par cas, sans appliquer systématiquement certaines solutions techniques, sauf à aller à l’encontre de l’objectif de rénovation. Il n’est ainsi pas souhaitable que la loi impose de recourir à certaines typologies de matériaux, car cela conduirait à rigidifier le dispositif. L’amendement n° 7 rectifié,

en établissant un diagnostic sérieux qui tienne mieux compte des particularités des collectivités d’outre mer et en émettant des recommandations de travaux également plus adaptées. Bien que l’échéancier soit différent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les logements classés G y seront interdits à la location au 1 janvier 2028, les logements classés F l’étant au 1 janvier 2031.

sur le fait que le DPE ne tient compte que des caractéristiques physiques du bâtiment, ce qui est un gage de fiabilité et de comparabilité. La performance énergétique du bâtiment ne peut reposer que sur des considérations physiques. Il n’est pas possible d’inclure d’inclure le climat dans le mode de calcul du DPE, sauf à le modifier, ce qui ne va pas dans le sens de la simplification. Sur le fond, j’ajoute que les apports de la commission permettent déjà de mieux prendre en considération ces conditions climatiques. En effet, les matériaux ont une empreinte locale forte. On ne retrouve pas les mêmes matériaux en Normandie, à Mayotte, en Guadeloupe et en Alsace ; ces derniers n’ont pas non plus les mêmes caractéristiques hygrothermiques. Or la commission a expressément précisé que les qualités hygrothermiques des matériaux des bâtis anciens, c’est à dire leur influence sur l’humidité et la température, seront prises en compte dans le cadre du DPE. J’estime que l’adoption de votre amendement

Je vous confirme, madame la sénatrice, que le Gouvernement a bien prévu d’adapter le DPE aux conditions climatiques particulières des départements et régions d’outre mer. d’outre mer. Cette adaptation s’impose du fait des dispositions inscrites au premier alinéa de l’article L. 126 26 du code de la construction et de l’habitation. En effet, en application de cet alinéa, le « diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment

objet de tenir compte également de leur perspirance et de leur inertie. En effet, respecter la perspirance et l’inertie thermique dans la rénovation des bâtiments anciens est essentiel pour éviter les pathologies du bâtiment, préserver ses caractéristiques architecturales et améliorer son confort thermique sans altérer ses qualités d’origine.

propose de prendre en compte l’hygrothermie lors des travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Comme je l’ai déjà expliqué, la prise en considération de la perspirance des matériaux utilisés pour l’isolation par l’extérieur est essentielle pour ne pas dégrader le bâti ancien. Si vous isolez par l’extérieur une maison à pans de bois avec du polystyrène,

chère collègue, s’inscrit dans un cadre très précis, celui du droit de surplomb du voisin en cas d’isolation thermique par l’extérieur. Je partage votre souci de favoriser des rénovations et des isolations respectueuses du bâti ancien. En revanche, je ne pense pas que la modification des règles relatives au droit de surplomb dans le cadre d’une isolation soit une manière pertinente de favoriser l’hygrothermie du bâti. À l’inverse,

que ce soit aux techniques employées ou aux matériaux utilisés. De plus, les rénovations énergétiques des bâtiments construits avec des techniques traditionnelles doivent déjà être respectueuses de ces bâtis et ne pas être à l’origine de pathologies futures, en particulier en garantissant une bonne ventilation – il s’agit de ne pas

rétablir une partie du dispositif de l’article 3 qui a été supprimée en commission des affaires économiques : il s’agit de préciser que le diagnostic de performance énergétique est également patrimonial.

ci tient également compte, par exemple, des contraintes techniques portant sur le bâti. Aussi, il paraît contre productif de complexifier la loi en introduisant cette référence au patrimoine dans l’intitulé

Par cet amendement, nous souhaitons interdire les isolations par l’extérieur sur des bâtiments qui ont des façades à pans de bois. En effet, les isolants synthétiques dérivés du pétrole, comme le polystyrène ou le polyuréthane,

cet amendement vont à l’encontre du compromis que nous avons adopté en commission. Je le rappelle, en 2025, les crédits budgétaires dédiés à MaPrimeRénov’ ont été réduits d’un milliard d’euros par rapport à 2024. En outre, les conditions actuelles d’octroi de la prime permettent déjà, dans certains cas, de réduire le reste à charge pour de lourdes rénovations du bâti ancien. Plutôt que de majorer systématiquement MaPrimeRénov’, nous proposons d’engager une réflexion sur les contours possibles d’un système de soutien spécifique à la rénovation énergétique des logements anciens qui éviterait tout effet d’aubaine,

Votre amendement, monsieur le sénateur, vise à instaurer une bonification de MaPrimeRénov’ pour les bâtiments anciens. Comme vous le savez, le contexte budgétaire est extrêmement contraint. Pour autant,

patrimonial, d’apposer une isolation à l’extérieur sur les façades. C’est pourquoi nous demandons l’extension du label de la Fondation du patrimoine aux travaux énergétiques à l’intérieur des bâtiments, lorsque ceux ci ne portent pas atteinte aux murs.

les objectifs de la Fondation du patrimoine vers la rénovation énergétique et entraînerait un saupoudrage des moyens. En outre, même s’il s’agit d’une recommandation de la commission d’enquête sur la rénovation énergétique, je constate que nous ne disposons pas d’évaluation chiffrée sur le montant de cette mesure, ce qui est dommage compte tenu du contexte budgétaire actuel.